Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, nous examinons aujourd’hui l’avenant à la convention entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale. Cette convention fiscale franco suisse, qui date du 9 septembre 1966, prévoit en règle générale que les revenus tirés d’un emploi salarié sont imposables au lieu d’exercice de l’activité. Cette disposition s’applique notamment aux travailleurs frontaliers qui résident en France et qui exercent une activité salariée dans le canton de Genève. Toutefois, l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des frontaliers français travaillant dans huit autres cantons suisses, que sont Berne, Soleure, Bâle Ville, Bâle Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura, dispose que ces revenus sont imposés dans l’État de résidence, c’est à dire en France. Cette spécificité s’explique par des raisons historiques. Le ministère d’Alsace Lorraine de l’Empire allemand et les cantons de Bâle Ville, Bâle Campagne et Soleure, par échange de lettres de 1910 et 1911, se sont entendus pour que les revenus des travailleurs frontaliers soient imposés uniquement dans leur État de résidence. Par succession de l’Allemagne en vertu du traité de Versailles, la France a repris ces engagements, qui ont été étendus par arrangement en 1935 à d’autres cantons. À la date de signature de ces accords, les migrations frontalières concernaient principalement des résidents suisses. En 1983, les parties sont convenues de maintenir la règle d’imposition en vigueur, alors même que le flux migratoire s’inversait. En contrepartie, elles se sont accordées sur le versement d’une compensation financière de 4,5 % de la masse totale des rémunérations brutes annuelles des travailleurs frontaliers par l’État de résidence à l’État du lieu de l’emploi. Par ailleurs, un accord du 29 janvier 1973 avec le canton de Genève prévoit que celui ci verse chaque année aux départements de l’Ain et de la Haute Savoie une compensation budgétaire non fiscale à hauteur de 3,5 % de la masse totale des salaires bruts des résidents en France travaillant dans ce canton. Cette somme vise à dédommager ces départements pour la charge liée aux infrastructures et aux services publics dont bénéficient ces frontaliers. Le montant de la compensation versée par le canton de Genève au titre de l’année 2023 s’est élevé à 372 millions de francs suisses, soit plus de 380 millions d’euros. Le présent avenant soumis à votre approbation s’inscrit dans la continuité du cadre juridique bilatéral en vigueur tout en le modernisant. Il a pour objectif d’encadrer l’activité du télétravail et d’appliquer à notre convention fiscale bilatérale les dernières normes internationales de l’OCDE pour la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, que nos deux États se sont engagés à respecter. L’essor du télétravail constaté lors de la crise du covid 19 a conduit les autorités françaises et suisses à neutraliser les effets du recours au télétravail sur le régime d’imposition des travailleurs frontaliers. Une succession d’accords amiables a été conclue en ce sens jusqu’en juin 2022 ; à compter de cette date, les administrations compétentes se sont accordées sur des règles d’imposition pérennes concernant l’exercice de l’activité en télétravail, formalisées dans deux accords amiables signés le 22 décembre 2022 et applicables à compter du 1 janvier 2023. Le présent avenant, signé le 27 juin 2023 à Paris, a pour objet d’inscrire dans la convention fiscale bilatérale les règles applicables au télétravail en dehors du cadre établi par l’accord de 1983 spécifique aux travailleurs frontaliers. Ainsi, à compter du 1 janvier 2023, les revenus issus de l’activité exercée en télétravail, dans la limite de 40 % du temps de travail annuel, restent imposables dans l’État où se situe l’employeur. En contrepartie, cet État verse à l’État de résidence du salarié une compensation financière fixée à 40 % des impôts dus sur ses rémunérations, étant précisé que, eu égard à la compensation budgétaire inscrite dans l’accord du 29 janvier 1973 intégralement préservée dans le cadre de cet accord, une règle de calcul spécifique s’applique lorsque l’employeur se situe dans le canton de Genève. Au delà de cette limite de 40 % du temps de travail, aucune compensation n’est due et le droit d’imposer les rémunérations correspondant à l’intégralité de la période télétravaillée revient à l’État de résidence du contribuable. S’agissant des frontaliers travaillant dans les huit cantons suisses précités, l’accord trouvé ne remet en cause ni le statut de frontalier ni les règles d’imposition à la résidence relevant de l’accord du 11 avril 1983. Ainsi, les revenus de ces travailleurs qui exercent leur activité en télétravail dans une limite de 40 % du temps de travail annuel demeurent imposables dans l’État de résidence. Au delà de cette limite, les règles de droit commun de la convention de 1966 s’appliquent. Le montant des compensations financières dues à raison de l’exercice du télétravail sera déterminé à partir des données accessibles par les administrations fiscales dans le cadre du nouveau dispositif d’échange de renseignements prévu à cet effet dans l’avenant. Ce dernier offre donc un cadre normatif fiscal novateur en matière de télétravail, équilibré pour nos finances publiques et adapté au contexte frontalier avec notre partenaire suisse son entrée en vigueur est très attendue par la communauté des frontaliers, estimée en 2024 à 230 000 travailleurs français, soit 58 % de l’ensemble des frontaliers en Suisse. Le texte soumis à votre approbation répond à un besoin de flexibilité concernant les modalités de travail, mais aussi de clarté des règles fiscales qui leur sont applicables. La multiplication du recours au télétravail dans ces conditions

Telles sont, monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu’appelle l’avenant à la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission des finances a examiné et adopté la semaine dernière ce projet de loi prévoyant l’entrée en vigueur d’un avenant à la convention fiscale franco suisse. Composé d’un article unique, ce texte a pour objet d’autoriser l’approbation de l’avenant du 27 juin 2023 modifiant la convention fiscale bilatérale du 9 septembre 1966. Comme vous le savez, en application de l’article 53 de la Constitution, l’entrée en vigueur de certains accords internationaux, dont les conventions fiscales, est subordonnée à l’autorisation du Parlement. Les projets de loi concernés, qui ne sauraient modifier le contenu des conventions, ont pour unique objet de valider ou de rejeter les solutions négociées par l’exécutif. Le Sénat se trouve être la première assemblée saisie de ce projet de loi, dont l’adoption par le Parlement est particulièrement attendue, l’avenant ayant été définitivement approuvé par un vote final de l’Assemblée fédérale suisse le 14 juin 2024. Sa mise en œuvre devrait affecter les plus de 236 000 personnes résidentes en France qui travaillent en Suisse. Revenons un instant sur les relations fiscales bilatérales entre la France et la Suisse. Cet encadrement repose non sur une seule convention fiscale bilatérale, comme il est d’usage, mais sur une série d’accords fiscaux et budgétaires qui établissent plusieurs régimes spécifiques. Cet enchevêtrement de textes découle de la répartition des compétences au sein de la Confédération helvétique et entre le niveau confédéral et les cantons. Deux accords principaux déterminent les relations fiscales bilatérales franco suisses.

Concernant l’imposition des travailleurs transfrontaliers, la convention retient à son article 17 un principe d’imposition dans l’État d’exercice de l’activité. C’est ce texte que vient modifier l’avenant qui fait l’objet de ce D’autre part, l’accord fiscal du 11 avril 1983 établit un régime frontalier entre la France et plusieurs cantons suisses. Les notions de travailleur frontalier et transfrontalier sont en effet distinctes. Un travailleur frontalier réside et travaille dans une zone frontalière définie par une convention bilatérale et se voit attacher un régime spécial. Par dérogation au principe du droit fiscal international, et contrairement à la convention de 1966, l’accord de 1983 retient un principe d’imposition dans l’État de résidence des rémunérations des travailleurs frontaliers. Il est applicable à huit cantons suisses : Berne, Soleure, Bâle Ville, Bâle Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. et Jura. Un accord spécifique en date du 29 janvier 1973, de nature budgétaire et non plus fiscale, concerne le seul canton de Genève, qui relève de la convention de 1966, et prévoit le versement aux deux départements frontaliers de ce canton, l’Ain et la Haute Savoie, d’une compensation financière équivalente à 3,5 % de la masse salariale brute des travailleurs transfrontaliers afin de financer les infrastructures qui bénéficient à ces derniers. Rappelons que plus de la moitié des transfrontaliers français en Suisse travaillent dans le canton de Genève, soit

a conduit à un fort développement du télétravail ; or son exercice a pour conséquence de modifier les modalités d’imposition pour les personnes résidant dans un État et travaillant habituellement pour un employeur situé dans l’autre État, l’État d’exercice de l’activité devenant l’État de résidence. Dans le but de neutraliser les effets fiscaux de l’essor du télétravail, la France et la Suisse ont conclu, à compter de 2020, une série d’accords amiables. En l’état du droit, deux accords en date du 22 décembre 2022 fixent les règles de partage d’imposition des activités effectuées en télétravail. Un premier accord traite de la situation des frontaliers relevant de l’accord de 1983 et dispose que l’exercice du télétravail dans la limite de 40 % du temps de travail ne remet en cause ni le statut de frontalier ni les règles d’imposition à la résidence des revenus d’activité salariée qui en découlent.

juin 2023. Un second accord concerne les transfrontaliers régis par la convention de 1966 et prévoit de maintenir l’imposition dans l’État de situation de l’employeur si le travail effectué à distance depuis l’État de résidence n’excède pas 40 % du temps de travail,

l’avenant de 1966 prévoit que l’État d’exercice de l’activité verse à l’État de résidence des télétravailleurs une compensation fiscale en contrepartie au renoncement par l’État de résidence à des recettes fiscales. Celle ci s’élève à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence. Un montant spécifique de compensation est prévu pour le canton de Genève afin de tenir compte des équilibres de l’accord budgétaire de 1973. l’adoption de cet avenant devrait renforcer la sécurité juridique des contribuables transfrontaliers et simplifier les règles applicables en matière d’imposition des rémunérations. Il contribuera également à désengorger le trafic routier entre la France et la Suisse, ce qui n’est pas négligeable. Toutefois, je tiens à tempérer cette appréciation par deux points d’attention. Premièrement, le Gouvernement n’a pas été en mesure de fournir une évaluation précise des conséquences de l’avenant pour nos recettes fiscales. La faiblesse de l’étude d’impact attachée au projet de loi est d’autant plus regrettable que la Cour des comptes, dans un référé de 2017, soulignait déjà l’insuffisance de l’expertise économique préalable à la négociation des conventions fiscales. Deuxièmement, l’application de l’avenant devra faire l’objet d’un suivi attentif quant à la mise en œuvre du mécanisme d’échange automatique d’information, prévue pour 2026, de la règle des dix jours de missions temporaires assimilables à du télétravail, qui suscite des inquiétudes chez certains travailleurs transfrontaliers. Le second volet de l’avenant de juin 2023 consiste en une mise à jour partielle de la convention de 1966 au dernier standard de l’OCDE. Le texte poursuit ainsi le travail de modernisation du réseau conventionnel français, à la fois au modèle de convention fiscale de l’OCDE mis à jour en 2017 et à l’instrument multilatéral de l’Organisation, issu du plan d’action pour lutter contre l’évitement fiscal et moderniser le droit fiscal international, mieux connu sous son acronyme anglais Beps L’avenant reprend les principales dispositions du modèle de convention de l’OCDE : il intègre une mise à jour du préambule de la convention au regard de l’objectif de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, une clause générale anti abus pour lutter contre certains montages fiscaux, une modernisation de la procédure de règlement des différends et un mécanisme d’ajustement corrélatif pour éviter les phénomènes de double imposition des bénéfices des entreprises.

l’accord trouvé entre la France et la Suisse me paraît équilibré et de nature à renforcer la sécurité juridique de nos contribuables transfrontaliers ainsi qu’à moderniser le cadre de nos relations fiscales bilatérales au regard des derniers standards internationaux.

de l’avenant du 27 juin 2023 à la convention franco suisse de 1966 et vous propose d’adopter le présent projet de loi sans le modifier. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, certaine rondeur diplomatique, chaque mot portant la trace des tractations patientes entre partenaires égaux, soucieux d’équilibre et de courtoisie, l’avenant qui nous est soumis engage une certaine conception de la justice fiscale et du partage de la valeur ajoutée entre nations. nations. Il révèle également une tension entre, d’une part, la nécessité d’une coopération entre administrations et la réalité d’une concurrence fiscale entre nos deux pays et, d’autre part, la transformation du travail lui même par de nouveaux modes d’organisation numérique. Pardonnez moi, mais il me semble que cet avenant cache un loup. Ce qui est en jeu, c’est une lente et méthodique érosion de notre capacité à décider des règles, celles d’un jeu fiscal au bénéfice d’un État qui, tout en affichant des gages de bonne volonté, demeure néanmoins, et très volontairement, l’un des derniers sanctuaires d’optimisation et d’évasion fiscales en Europe. C’est là toute l’utilité pour la Suisse des avenants signés avec la France dans les années 2000 2010. L’objectif était de sortir de la liste noire, puis de la liste grise des paradis fiscaux en 2019,

Au demeurant, cet avenant fait l’impasse sur la matrice des stratégies de domiciliation artificielle des profits et de l’imposition effective des flux financiers offshore, mais prétend instaurer un nouveau partage de la fiscalité sur le télétravail des frontaliers. Or nous constatons que l’État helvétique en ressort triplement gagnant.

deuxièmement, il capte une part significative de la valeur ajoutée produite par ces salariés. Pourtant, les charges collectives qui leur sont associées reposent largement sur la France. Ces travailleurs sont formés dans notre système éducatif, logés sur notre territoire et bénéficient de nos infrastructures, routes, transports, crèches, hôpitaux, connexions, fibre. Qui plus est, selon les données de l’Urssaf, 68 % d’entre eux sont affiliés à la sécurité sociale française.

même : « Les cantons et les milieux économiques concernés ont accueilli favorablement la conclusion de l’avenant. » Le rapporteur suisse du texte ajoute : « Cette solution est très favorable à la Suisse et meilleure que celle négociée avec l’Italie. »

Bercy consent à une fiscalité en berne et à une convention profondément déséquilibrée ! Pour autant, le problème est encore plus vaste. Cette mesure engendre un effet d’aubaine : tous les cadres salariés chercheront naturellement à maximiser leur télétravail sous le seuil fixé à 40 40 %, avec la complicité tacite des employeurs suisses. Autrement dit, nous laissons libre cours aux optimisations discrètes et aux arrangements officieux. Cette doctrine fiscale est d’une complaisance inquiétante, alors que

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, depuis la crise sanitaire, le télétravail s’est imposé dans nos quotidiens, bouleversant nos habitudes et redéfinissant nos relations économiques. Comme pour un mécanisme d’horlogerie, chaque ajustement à cette évolution structurelle doit être opéré avec précision et mesure. Il s’agit ici de garantir une coopération fiscale franco suisse mieux équilibrée, tout en évitant la double imposition et l’évasion fiscale. Première terre d’accueil de nos compatriotes à l’étranger et partenaire commercial essentiel, la Suisse entretient avec la France des liens étroits et historiques. Face à une hausse de 19 % du nombre des frontaliers en seulement quatre l’encadrement du télétravail est une nécessité. L’intégration du pilier 2 de l’OCDE dans le cadre de la réglementation Beps marque à cet égard une étape importante.

comment mesurer ses effets réels sur l’emploi frontalier et ses conséquences économiques et fiscales ? La Cour des comptes a déjà soulevé cette critique dans son référé de mai 2019 sur les conventions fiscales internationales, relevant que l’expertise économique préalable aux négociations était insuffisante et que les moyens consacrés au suivi des conventions fiscales devaient être renforcés. Ensuite, l’avenant prévoit un ajustement corrélatif des prix de transfert entre entreprises associées. Quels mécanismes concrets permettront cependant de prévenir les risques de pratiques d’optimisation fiscale ? de régulation stricte, certaines entreprises pourraient déplacer leurs bénéfices vers la Suisse, où le taux minimal de 15 % imposé par l’OCDE aux grandes entreprises dans le cadre de cette convention reste inférieur au taux de 25 % appliqué en France. Enfin, un autre déséquilibre est mis en lumière. Alors que les travailleurs transfrontaliers profitent d’une fiscalité plus avantageuse en Suisse, une partie des coûts sociaux qu’ils engendrent repose sur les finances publiques françaises. En Suisse, le salaire moyen atteint 4 382 euros nets, contre 2 735 euros en France. Lorsque ces travailleurs perdent leur emploi, ils perçoivent des allocations chômage suisses calculées sur leur salaire pour une durée de trois à cinq mois avant de basculer sur le régime français. Ce transfert de charges assumé par les entreprises françaises pèse lourdement sur l’Unédic et fragilise le financement de France Travail, avec des pertes estimées à plusieurs milliards d’euros. Une convergence entre nos deux pays sera nécessaire pour garantir un cadre financier plus équilibré. Malgré ces écueils certains, et alors que les discussions entre la France et la Suisse semblent être définitivement au point mort sur la nouvelle convention fiscale en matière de succession, cet avenant à la convention fiscale franco suisse en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est utile. Même s’il reste partiel, il constitue une avancée notable vers une coopération fiscale plus adaptée aux réalités de nos citoyens frontaliers. En conséquence, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera en faveur de ce texte. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui un projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention fiscale entre la France et la Suisse, un texte qui un texte qui recèle des enjeux concrets pour des milliers de travailleurs frontaliers et pour nos finances publiques. En tant que sénatrice de l’Ain, je suis particulièrement attentive à cette question. Mon département comporte une forte proportion

au profit de l’État de résidence des transfrontaliers télétravailleurs lorsque le travail à distance excède 40 %. Ce versement de 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées

qu’en 2026, retardant l’application effective de ce mécanisme. En outre, l’avenant prévoit que les missions temporaires exercées par un salarié dans son État de résidence ou dans un pays tiers, lesquelles sont fréquentes, sont assimilées à du télétravail,

affirmant explicitement l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale ; il introduit une clause anti abus pour éviter les montages fiscaux ayant un objectif principalement fiscal ; il réforme le règlement des différends, en permettant à toute personne estimant subir une imposition non conforme de saisir l’une ou l’autre des administrations fiscales compétentes ; et il prévoit un ajustement corrélatif pour éviter la double imposition liée aux prix de transfert.

pas moins une avancée. Il permet d’adapter notre cadre fiscal aux réalités du travail transfrontalier tout en renforçant, au moins en principe, les outils de lutte contre l’évasion fiscale. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera

une histoire européenne, un attachement à la démocratie libérale et une coopération transfrontalière dynamique. C’est ainsi que 200 000 Suisses résident de manière pérenne en France et que 200 000 Français vivent dans les cantons suisses. En sus de ces importantes populations d’expatriés, 200 000 Suisses traversent chaque jour la frontière pour venir travailler en France, pendant que 220 000 Français font le chemin inverse pour aller exercer leur Au total, ce sont 800 000 nationaux de nos deux pays qui vivent de cette relation singulière entretenue par la Suisse et la France. Les liens noués avec cet État non membre de l’Union européenne sont donc très forts, à l’instar de ceux qui nous unissent au Royaume Uni.

La Suisse, qui est parfois décrite comme un paradis fiscal, est surtout un pays qui parvient à offrir à sa population un très haut niveau de services publics tout en ayant une fiscalité particulièrement faible. Sa productivité, son excellente industrie et sa fiscalité en font un îlot au milieu de l’Union européenne dont nous ferions bien de nous inspirer. La Suisse est le troisième pays de l’OCDE en matière de niveau de vie de ses habitants, quand la France n’est classée qu’au neuvième rang. Le patrimoine net moyen des ménages est près de deux fois supérieur en Suisse qu’en France. Quant au salaire moyen, il s’élève à 2 300 euros dans notre pays, contre 7 000 euros chez notre voisin, qui connaît en outre un taux de chômage très faible de 2,9 %, contre plus de 7 % en France. Les habitants des territoires frontaliers sont donc inévitablement attirés à l’idée d’aller travailler en Suisse. Nos concitoyens de Haute Savoie, du Haut Rhin, du Doubs, de l’Ain, du Jura et du Territoire de Belfort sont chaque année toujours plus nombreux à traverser la frontière pour rejoindre leur lieu de travail. Depuis 2010, leur nombre a ainsi augmenté de 86 %. Cette disparité entre nos deux pays conduit tout de même, il faut le signaler, à vider une partie de nos départements de leur main d’œuvre. Les employeurs français des départements concernés ne peuvent absolument pas aligner les salaires qu’ils proposent sur ceux qui sont promis en pays helvète.

Pour permettre aux populations locales de continuer à vivre dans la commune, les élus ont été obligés d’imposer un encadrement des loyers dont chacun sait qu’il ne constitue pas la solution idéale. Comme nos deux pays partagent, si je puis dire, une partie de leurs travailleurs, il a fallu signer des conventions afin de régler les modalités d’imposition. Tel est l’objet des conventions de 1966 et de 1983, que l’avenant soumis à notre examen aujourd’hui met à jour met à jour s’agissant du régime des télétravailleurs, notamment des résidents français qui, travaillant habituellement de l’autre côté de la frontière, exercent en partie leur métier depuis notre territoire. Afin d’éviter tout abus,

cotisent pour le chômage en Suisse, à raison des salaires très élevés qu’ils perçoivent, tout en étant indemnisés par la France le jour où ils se retrouvent sans emploi. La disparité de revenus entre nos deux pays et les règles de licenciement, beaucoup plus souples en Suisse qu’en France, sont à l’origine du déficit particulièrement important que nous subissons chaque année.

de revenus. Notre groupe votera ce projet de loi, mais nous appelons avec beaucoup d’insistance à revoir les relations sociales qui nous lient avec les pays frontaliers, en particulier avec nos amis suisses. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui vise à autoriser l’approbation de l’avenant à la convention fiscale franco suisse. Cette convention régit notamment l’imposition de 220 000 résidents français travaillant en Suisse, dont plus de 110 000 personnes dans le seul canton de Genève. Le principe est l’imposition dans l’État d’exercice de l’activité salariale, avec des exceptions pour certains cantons. ce dispositif conventionnel fonctionne bien, le présent avenant permettra de moderniser notre cadre bilatéral en prenant acte des mutations profondes de notre marché du travail. Cet avenant établit un nouveau régime d’imposition du télétravail frontalier.

En contrepartie, l’État employeur verse à l’État de résidence une compensation fiscale équivalente à 40 % du montant de l’imposition des rémunérations

Au delà du télétravail, l’avenant intègre également une clause anti abus conforme au modèle de l’OCDE et met en œuvre un échange automatique de données fiscales qui sera pleinement opérationnel en 2026. Ce texte est donc à la fois pragmatique pour les travailleurs et équilibré pour les États. Sa mise en application devra toutefois être suivie avec beaucoup de vigilance. Trois interrogations subsistent en effet. La première a trait au seuil des dix jours de missions temporaires assimilables au télétravail.

au manque de visibilité relative au montant des compensations futures. La signature d’une convention ou d’un avenant ne garantit pas à elle seule la sécurité juridique et fiscale. L’exemple italien montre que cette sécurité fiscale tient non pas seulement à la lettre d’un traité, mais à sa mise en œuvre cohérente, bilatérale, transparente et pérenne. pérenne. Jusqu’en 2021, les Français résidant en Italie et percevant une pension relevant du régime général de la sécurité sociale étaient uniquement imposés en France. Subitement, pour des raisons que l’on ne connaît pas, à la suite d’un changement d’interprétation par l’administration fiscale italienne, ces résidents français vivant en Italie, retraités et professeurs, se sont vus réclamer des impôts sur leur retraite ou sur leur rémunération en plus de leur imposition française, assortie de sanctions et d’intérêts exorbitants, et ce rétroactivement, à compter de 2015. de 2015. Un manque de vigilance dans la mise en œuvre d’une convention peut emporter des dettes fiscales s’élevant à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euros. Certains ont dû vendre leur logement, d’autres ont tout perdu.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est essentiel pour moderniser notre cadre fiscal avec la Suisse. Il actualise la convention de 1966 afin de clarifier les règles d’imposition applicables aux plus de 236 000 travailleurs transfrontaliers, tout en pérennisant un système fiscal équilibré et en assurant une répartition équitable des recettes entre nos deux pays. contribuera également à renforcer la lutte contre la fraude fiscale, un enjeu particulièrement cher à notre assemblée, comme l’ont illustré nos débats d’hier soir.

Il introduit une clause anti abus afin de contrer les montages fiscaux artificiels et élargit les possibilités de recours en cas de différend – tout un chacun pourra ainsi saisir les autorités compétentes en cas de suspicion d’imposition non conforme à la convention. Cet avenant contribuera également à pérenniser les accords temporaires relatifs au télétravail qui ont été conclus durant la crise du covid 19. Sans cadre adapté, les salariés travaillant à distance risquaient de voir leurs règles d’imposition bouleversées. Désormais, jusqu’à 40 % du temps de travail pourra être effectué à distance sans remettre en cause les règles d’imposition à la résidence des revenus d’activité salariée. L’avenant à la convention de 1966 va toutefois plus loin, car il introduit une compensation fiscale au profit de l’État de résidence des transfrontaliers télétravailleurs. Nous devons nous en féliciter, car la France devrait bénéficier de cette

Comme plusieurs de mes collègues, je m’inquiète également de la fixation à dix jours de la durée maximale des missions temporaires assimilables à du télétravail. De nombreux transfrontaliers, notamment en raison de la forte présence d’organisations internationales en Suisse, doivent effectuer des déplacements fréquents. Cette mesure pourrait donc poser de nouvelles difficultés.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au moment où nous discutons de ce projet de loi, 230 000 travailleurs français traversent chaque jour la frontière suisse pour travailler, soit 86 % de plus qu’en 2010. Permettez moi de rappeler, en préambule, que si la Constitution limite les prérogatives de notre Parlement en matière de relations internationales, son rôle n’en est pas moins important. l’avenant en discussion aujourd’hui aurait dû être ratifié en 2024, puis entrer en vigueur en 2025, mais les perturbations politiques survenues en 2024, dont la nature doit sembler bien exotique à nos voisins helvètes, en ont décidé autrement. Dans l’urgence, les accords amiables conclus en 2020 ont permis d’apporter une première réponse temporaire pour neutraliser les effets de bord fiscaux. La signature du présent avenant n’en était pas moins essentielle, non seulement pour clarifier le droit applicable, mais aussi pour statuer sur la question sensible de la compensation financière.

bilatérale franco luxembourgeoise, qui a rétabli des règles fiscales plus équitables. L’avenant que nous examinons aujourd’hui obligera les cantons suisses concernés, à l’exception de celui de Genève, à effectuer un versement à hauteur de 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis la France. Pour le canton de Genève, cette compensation ne concernera que la fraction de télétravail comprise entre 15 % et 40 % de télétravail par an. Quel sera le le montant de cette compensation pour la France ? Et surtout, quels seront les effets de ces nouvelles règles pour les contribuables français concernés ? Personne ne sait répondre à ces questions aujourd’hui, pas même l’administration fiscale, qui a produit une étude d’impact lacunaire sur les conséquences de cet avenant.

soulève des préoccupations chez nos travailleurs français établis en Suisse. Ma collègue Sophie Briante Guillemont a été alertée sur les risques de requalification fiscale abusive et sur le climat d’insécurité juridique que cette disposition pourrait emporter. J’appelle donc l’administration fiscale française à traiter ces sujets avec la plus grande attention. Enfin, l’examen de ce projet de loi permet de mettre une nouvelle fois en lumière le coût qu’emporte l’assurance chômage des travailleurs transfrontaliers.

permettez moi de saluer le travail remarquable accompli par notre collègue Sylvie Vermeillet en sa qualité de rapporteure du présent projet de loi.

Comme vous le savez, l’article 53 de notre Constitution exige que certains accords internationaux, en particulier les conventions fiscales, soient autorisés par le Parlement. Sans modifier le contenu des négociations conduites par l’exécutif, nous décidons donc simplement d’en entériner ou d’en refuser les conclusions. Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui a pour visée d’autoriser l’approbation de l’avenant du 27 juin 2023 modifiant la convention fiscale franco suisse du 9 septembre 1966. Les règles de partage de l’imposition des travailleurs transfrontaliers entre la France et la Suisse sont aujourd’hui déterminées par deux accords principaux – cela a été rappelé à maintes reprises depuis le début de nos débats. est la convention fiscale du 9 septembre 1966, dont il est principalement question aujourd’hui, qui établit comme principe l’imposition dans l’État d’exercice de l’activité. Le second est l’accord du 11 avril 1983,

des transfrontaliers entre les deux pays. Afin de clarifier l’incidence fiscale du télétravail et d’en neutraliser les effets indésirables, les autorités françaises et suisses ont conclu dès 2020 des accords fiscaux amiables. Un premier accord, applicable aux frontaliers relevant de l’accord de 1983, stipule que l’exercice du télétravail, dans la limite de 40 % du temps de travail, ne remet pas en cause les règles d’imposition. Un second accord, applicable aux travailleurs relevant la convention de 1966, maintient l’imposition dans l’État de l’employeur lorsque le télétravail n’excède pas 40 % du temps de travail, tout en prévoyant l’imposition dans l’État d’exercice de l’activité lorsque ce seuil est dépassé.

net – s’élevant à 40 % des impôts dus sur les rémunérations versées à raison des activités exercées en télétravail depuis l’État de résidence. de résidence. L’avenant participe ainsi d’une simplification administrative souhaitée par les employeurs comme par les salariés tout en renforçant la sécurité juridique du régime du télétravail transfrontalier. Le second volet modernise la convention de 1966 en l’alignant sur les derniers standards de l’OCDE. L’avenant intègre à cet effet les dernières avancées en matière de lutte contre les pratiques d’optimisation et de fraude fiscales. Il prévoit notamment la mise à jour du préambule de la convention au regard des objectifs de lutte contre les fraudes, l’intégration d’une clause anti abus pour lutter contre les montages fiscaux abusifs, l’élargissement des possibilités de saisine des contribuables en cas de différends fiscaux ou encore l’introduction d’un mécanisme d’ajustement pour éviter les phénomènes de double imposition. intègre en outre à la convention de 1966 un nouvel article qui garantit l’applicabilité des règles du pilier 2 de l’OCDE relatives à l’imposition minimale des entreprises. Quelques points de vigilance soulevés par notre rapporteur doivent retenir toute notre attention, mes chers collègues. Il est regrettable que le Gouvernement n’ait pas été en mesure de fournir une évaluation précise des conséquences précise des conséquences de l’avenant sur nos recettes fiscales, ce qui fragilise l’appréciation financière de ce texte. L’échange automatique d’informations prévues pour 2026

de convention de l’OCDE. Cet avenant apporte toutefois des ajustements nécessaires au renforcement de la sécurité juridique des contribuables transfrontaliers et à la modernisation du cadre de nos relations fiscales bilatérales.

La séance est suspendue. La séance est reprise. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte

a pour objectif d’apporter une première réponse à cette situation qui pèse sur l’économie locale et sur le fonctionnement des services publics. publics. Le dispositif proposé prévoit à cette fin de restreindre les possibilités d’acquisition de la nationalité française, sur le seul territoire mahorais, par le biais du droit du sol, en aggravant la première dérogation introduite en 2018. Nous examinons aujourd’hui le texte de compromis résultant des travaux de la commission mixte paritaire, qui conserve une partie des apports du Sénat. Nous nous étions en particulier attachés, en commission comme en séance publique, à sécuriser juridiquement le dispositif proposé afin d’éviter toute censure du Conseil constitutionnel. Je me félicite en premier lieu du maintien de la durée d’un an de séjour régulier en France, introduite par le Sénat. Le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire prévoit ainsi qu’un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne pourra devenir français au titre du droit du sol que si ses parents résident régulièrement en France depuis au moins un an à sa date de naissance.

permettant de ne pas priver un enfant né à Mayotte et issu d’une famille monoparentale de la possibilité d’accéder ultérieurement à la nationalité française. Je considère que la rédaction que nous avons retenue est pleinement satisfaisante et permettra de rendre la disposition plus dissuasive, en limitant les possibilités de fraude, tout en conservant son caractère proportionné. Enfin, la commission mixte paritaire a souhaité rétablir l’obligation pour les parents de présenter un passeport biométrique à l’officier d’état civil, pour apposer, sur l’acte de naissance de l’enfant, une mention relative à leur durée de séjour régulier en France. L’objectif est de lutter contre la fraude documentaire à Mayotte, qui constitue une voie de contournement de la restriction au droit du sol que nous introduisons en parallèle. Si cette intention est louable et si je suis satisfait du compromis trouvé,

Il s’agit toutefois d’un premier pas pour tenter d’endiguer les flux migratoires irréguliers constatés sur l’île. En attendant la mobilisation d’autres leviers, je vous invite, mes chers collègues, à adopter le texte issu des travaux de la commission mixte

que connaissent nos compatriotes mahorais depuis le mois de décembre dernier, quand l’archipel a été ravagé par le cyclone Chido. Je défendais alors la volonté du Gouvernement, sous l’autorité du Premier ministre, de s’attaquer aux urgences vitales, puis de préparer la reconstruction, avant d’entamer la refondation.

le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte, ainsi qu’un projet de loi organique qui aura vocation à « réarmer » la collectivité de Mayotte. Ces deux textes, que vous examinerez avant le mois de juin prochain, sont – je le crois – à la hauteur des attentes des habitants de Mayotte et des élus mahorais. Et je sais pouvoir compter sur les parlementaires pour les enrichir. Je vous le disais au moment de l’examen du projet de loi d’urgence, « si le cyclone a ravagé Mayotte, il a surtout révélé et exacerbé des calamités qui existaient déjà, un sous développement des infrastructures économiques et des services publics, entretenu par deux fléaux qui rongent l’île depuis des années : l’habitat illégal et l’immigration clandestine Mesdames, messieurs les sénateurs, il nous faut éviter, après les réponses exceptionnelles que nous avons apportées à la catastrophe qu’a traversée Mayotte, de revenir à la situation antérieure, sans rien changer aux problèmes du passé.

aussi ce que prévoit la présente proposition de loi, qui vise à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte et qui a fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire auquel le Gouvernement souscrit pleinement. Mayotte n’est pas un territoire comme un autre. C’est le plus jeune département de la République ; c’est aussi celui où l’écart est le plus grand entre les principes de notre droit et les réalités démographiques, sociales et migratoires. Sur ce territoire, près d’un habitant sur deux est de nationalité étrangère. Chaque année, plus de 10 000 enfants y naissent, soit vingt cinq par jour, dans des conditions souvent précaires et parfois dramatiques. Près de trois quarts d’entre eux ont une mère en situation irrégulière. Chaque année, des milliers de femmes enceintes traversent l’océan, bravant tous les dangers, souvent au péril de leur vie, pour accoucher sur le territoire, animées par l’espoir que ces naissances ouvriront un jour la voie à une régularisation et à une naturalisation.

Cette situation a des conséquences dramatiques sur la vie de nos compatriotes mahorais et sur le fonctionnement de l’État : les écoles sont surchargées, avec des classes de plus de cinquante élèves se partageant parfois une seule salle, sans maîtrise suffisante du français et sans aucune condition d’apprentissage digne le système de santé est complètement saturé – je pense en particulier à la maternité qui accueille, en majorité, des femmes sans titre de séjour ; l’insécurité ronge l’île, avec un taux de délinquance élevé, des tensions communautaires croissantes et des violences urbaines régulières ; plus récemment, le cyclone Chido a mis à rude épreuve la cohésion sociale et mis encore davantage en exergue les fragilités du territoire. Face à cette situation, l’État n’a pas reculé. Depuis 2017, les effectifs de police et de gendarmerie ont doublé. En 2023, plus de 25 000 reconduites à la frontière ont été effectuées à Mayotte, soit un tiers des expulsions prononcées sur l’ensemble du territoire national. Nous devons cependant le reconnaître : la seule réponse administrative ou répressive ne suffira pas.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la proposition de loi présentée par le député Philippe Gosselin. Je veux saluer ici la constance de son engagement sur cette question, tout comme celle du rapporteur pour le Sénat, Stéphane Le Rudulier. de loi vise à adapter notre droit de la nationalité aux spécificités de Mayotte, dans le respect du cadre constitutionnel et des exigences de l’État de droit. Le texte issu de la commission mixte paritaire introduit trois modifications majeures. mois à un an de la durée de résidence régulière requise pour les parents. Cette durée est raisonnable, proportionnée et juridiquement défendable : elle permet de limiter les accouchements de circonstance, qui visent moins à protéger l’enfant qu’à créer un ancrage administratif pour l’ensemble de la famille. loi l’exigence de résidence régulière des deux parents, lorsqu’ils sont tous deux identifiés comme tels. Cette précision est fondamentale, car elle permettra de lutter contre les reconnaissances frauduleuses de paternité, souvent organisées en échange d’une somme d’argent, et qui visent à contourner les règles d’accès à la nationalité.

Je le dis avec gravité : ce texte ne remet pas en cause le droit du sol – ce serait contraire à notre Constitution –, mais il en encadre strictement les effets, par souci de cohérence et d’équité. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 septembre 2018, a expressément reconnu que des adaptations spécifiques peuvent être apportées à Mayotte, dès lors qu’elles sont justifiées, limitées et proportionnées. C’est bien le cas ici. Mesdames, messieurs les sénateurs, ce texte est une réponse attendue, nécessaire, juste. Il permet à la République de parler un langage clair, adapté, exigeant. Il renforce la cohésion sociale à Mayotte. Il garantit que l’accès à la nationalité repose désormais sur une présence réelle, régulière et sincère sur notre sol. C’est pourquoi, au nom du Gouvernement, je vous invite à adopter sans réserve les conclusions de la commission mixte paritaire. texte ne permettra pas de relever tous les défis de Mayotte, mais il apporte une réponse structurante, solide et conforme à nos valeurs. Surtout, il envoie un message clair à nos compatriotes mahorais : la République est là ; elle écoute ; elle agit

Mahorais. Ernest Lavisse, cet historien républicain qui a inspiré des générations de hussard noirs et d’écoliers, nous rappelait une vérité essentielle : on apprend à être Français. Être Français, ce n’est pas un héritage figé, inscrit dans le marbre du sang ou du sol, c’est une construction éducative, culturelle, une volonté d’appartenance partagée. Or nous sommes aujourd’hui réunis pour examiner les conclusions de la commission mixte paritaire sur une proposition de loi en totale contradiction avec cet idéal républicain. Ce texte, inspiré par l’extrême droite, défendu par la droite et soutenu par le camp gouvernemental ouvre une nouvelle brèche dans notre pacte républicain. Il restreint encore davantage les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte, sous couvert de pression migratoire. Mayotte traverse une crise sans précédent. Après le passage du cyclone Chido, à l’origine de destructions majeures, les Mahorais attendaient une réponse forte de l’État. Ils espéraient un engagement concret pour reconstruire, améliorer leurs conditions de vie, renforcer leurs infrastructures. Au lieu de cela, quelle réponse leur apporte t Un débat nauséabond sur le droit du sol, instrumentalisé par ceux qui refusent d’assumer leurs responsabilités. La présente proposition de loi renforce un régime dérogatoire spécifique à Mayotte en allongeant la durée de résidence régulière exigée des parents d’un enfant né sur le territoire. Désormais, ce ne sera plus trois mois, mais un an ! Désormais, ce ne sera plus un seul parent, mais les deux ! Ce durcissement n’apporte aucune solution aux véritables problèmes de Mayotte ; il ne fait que désigner un bouc émissaire : l’étranger !

Un tiers des habitants n’avaient pas accès à l’eau potable. Les infrastructures publiques étaient sous dimensionnées. Les trois quarts de la population vivaient sous le seuil de pauvreté. Comment peut on, dans ces conditions, faire croire que la solution passe par la restriction du droit du sol ? La vérité, c’est que l’État a failli. En laissant Mayotte dans une précarité indigne, en refusant d’investir à la hauteur des besoins, en traitant ce département comme une périphérie lointaine plutôt que comme une partie intégrante de la République. Mayotte mérite mieux que cela. Elle mérite des écoles dignes de ce nom, des hôpitaux modernes, des infrastructures adaptées. Elle mérite aussi l’égalité réelle, et non une législation d’exception qui la stigmatise encore davantage… L’urgence est aussi climatique et nous n’y répondrons ni par le droit du sol ni par des barrières, mais par des politiques visionnaires et des infrastructures adaptées. La nature ne connaît pas de frontières : les cyclones ne s’arrêtent pas aux lignes tracées sur une carte ; la montée des eaux ne distingue ni nationalité ni statut administratif. À Mayotte comme ailleurs, c’est l’inaction qui aggrave les vulnérabilités. Plutôt que de dresser des murs, investissons dans des solutions durables protection du littoral, accès à l’eau potable, transition énergétique. Sans cela, nous ne ferons que subir, impuissants, les catastrophes à venir. Comprenons bien une chose : nous ne relèverons pas les défis migratoires de Mayotte en fermant les yeux sur leur origine profonde. La pression migratoire existe, c’est un fait. Mais comment peut on sérieusement prétendre y répondre, alors que nous avons réduit de 37 % Comment peut on prétendre stabiliser cette région sans une politique ambitieuse de codéveloppement ? Car la réduction de 37 % du budget consacré à l’aide au développement ne fait qu’aggraver les migrations forcées. Au delà des chiffres, c’est notre incapacité à changer de paradigme dans notre relation avec l’Afrique qui nourrit cette dynamique migratoire. Tant que nous continuerons à voir ce continent uniquement à travers le prisme de l’urgence sécuritaire et migratoire, nous ne ferons que repousser les solutions nécessaires à un avenir plus stable et partagé. Aimé Césaire nous mettait en garde : « Une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. » Sommes nous prêts à voir la République renier renier ses principes fondamentaux au nom du repli identitaire ? Sommes nous prêts à abandonner nos compatriotes mahorais à une pauvreté structurelle, tout en leur désignant l’étranger comme coupable de tous leurs maux ? Mayotte nous rappelle une chose essentielle : nous ne pouvons pas laisser se perpétuer une République à deux vitesses ! Nous ne pouvons pas accepter que nos territoires ultramarins soient relégués au rang de « sous France » ! Nous devons au contraire leur offrir une égalité réelle, leur consacrer des investissements à la hauteur et une attention sincère. Car Mayotte n’est pas un simple territoire lointain, c’est une partie de notre République ! Ses habitants demandent non pas la charité, mais la justice ! Ils demandent à vivre dignement, comme n’importe quel citoyen français. Il est temps de répondre à cet appel, non par des lois qui excluent, mais par des politiques qui intègrent. Vous l’aurez compris, nous ne voterons pas ce texte. La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous apprêtons à entériner une nouvelle entaille dans un principe fondamental de notre République : le droit du sol. Vous choisissez de vous attaquer à l’indivisibilité de notre République, après l’avoir déjà fait une première fois en 2018 avec la loi Asile et Immigration. En effet, depuis plus de six ans, il faut, pour qu’un enfant devienne français à Mayotte, qu’au moins l’un de ses parents ait résidé sur le territoire mahorais de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Vous nous proposez une nouvelle fois de modifier la loi, alors qu’aucune évaluation de la loi de 2018

a été multiplié par dix et le nombre de naissances sur l’île n’a cessé d’augmenter, en hausse de 47 % entre 2014 et 2022. Nous savons également que la réforme de 2018 n’a fait qu’accroître la grande précarité de nombreuses familles et de jeunes, privés d’accès à la nationalité française et obligés de survivre sur le territoire. Les débats autour de cette proposition de loi nous ont contraints à écouter les arguments et les fantasmes les plus nauséabonds sur l’immigration : l’idée que les migrants se livreraient à un, pèseraient le pour et le contre d’une traversée sur un kwassa kwassa en risquant leur vie, afin d’être certains que leurs enfants pourront bénéficier de la nationalité française l’idée que les femmes ne sont finalement que des « ventres » destinés à faire des enfants et qu’elles viendraient cyniquement accoucher sur des plages à Mayotte, les ramenant à leur condition la plus animale. la plus animale. C’est tellement plus facile de ne pas se demander quelles considérations sociales, économiques ou politiques les poussent à fuir la misère et, parfois, la mort. tellement plus facile de ne pas vouloir investir financièrement dans les services publics et les infrastructures à Mayotte. C’est tellement plus facile d’ignorer la nécessité de politiques de coopération d’ampleur avec les Comores. Assurément, réformer le droit du sol et s’attaquer à l’étranger coûte bien moins cher

En huit ans, nous n’allons pas vous apprendre que la situation s’est aggravée et que les tensions se sont exacerbées… Comme en première lecture, nous sommes fermement opposés à ce texte. Chose assez rare pour être soulignée, la commission mixte paritaire a durci la version du Sénat,

ailleurs, la rédaction retenue par la commission mixte paritaire pour définir les familles monoparentales risque fortement d’entraîner des non reconnaissances d’enfants et de créer des situations très dangereuses. Je l’ai dit lors de la réunion de la CMP : la monoparentalité ne tient pas seulement à la déclaration de filiation à la naissance, car l’un des parents peut décéder très peu de temps après la naissance ou avoir déserté. La question du non respect de l’égalité des enfants devant la loi reste entière. Cette mesure fait peser un risque d’inconstitutionnalité sur le texte. Finalement, l’atteinte manifeste et disproportionnée de cette proposition de loi au droit du sol n’est ni justifiée ni adaptée. Il n’a jamais été démontré depuis 2018 que la réforme du droit du sol avait endigué les flux migratoires. de mettre un pied dans la porte pour remettre en cause le droit du sol sur tout le territoire français, ce à quoi même le régime de Vichy n’avait pas osé toucher Nous, sénateurs socialistes, continuerons de nous opposer jusqu’au bout à ce texte inutile, populiste et xénophobe. Nous saisirons le Conseil constitutionnel pour Mayotte et pour tous ces enfants qui méritent bien mieux

Prise au piège d’un poids démographique devenu insoutenable, soumise à des flux migratoires continus, avec comme corollaire la saturation des services publics, l’explosion de l’insécurité, l’insalubrité des habitats ou encore la dégradation de l’environnement, Mayotte est en train de sombrer. Ce département français de l’océan Indien subit, depuis de trop longues années, un détournement systématisé du droit du sol, utilisé comme un outil d’ingérence par un pays étranger contestant la souveraineté de la France sur l’archipel. Revendiquant l’appartenance de Mayotte à son territoire, malgré plusieurs référendums confirmant le souhait des Mahorais de rester au sein de la République française, l’Union des Comores instrumentalise les flux migratoires à des fins de déstabilisation et de prise de contrôle. Face à une catastrophe migratoire d’une telle ampleur, il est de notre responsabilité de protéger notre territoire, afin d’assurer la sécurité de nos concitoyens. Pour cela, une gestion responsable de l’immigration s’impose.

Certes, elle n’est pas parfaite et ne réglera pas tout, mais nous posons une première pierre en envoyant un signal fort : les Mahorais ne sont pas seuls pour affronter les défis immenses posés par cette immigration hors de contrôle. Ce texte a le mérite de restaurer une forme d’équilibre en alignant le droit sur les réalités démographiques et sociales de Mayotte. C’est pourquoi je me félicite de l’esprit consensuel qui a prévalu lors de la réunion de la commission mixte paritaire, qui a permis d’aboutir à un accord pour adapter les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte. Je me réjouis tout particulièrement que ce soit la version du Sénat, qui fixe à un an la durée de résidence régulière exigée des parents à la date de naissance de l’enfant, afin qu’il puisse accéder ensuite

Enfin, je suis favorable à l’obligation de présentation d’un passeport biométrique pour apposer sur l’acte de naissance de l’enfant la mention de la durée de la résidence régulière en France de ses parents. Avant de conclure, je tiens à remercier le rapporteur, notre collègue Stéphane Le Rudulier, de son travail remarquable et de son implication. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l’immigration irrégulière est un fléau à Mayotte. Elle porte atteinte à nos valeurs républicaines.

Il semble tout aussi urgent d’agir par la voie diplomatique, dans le cadre de nos relations bilatérales avec l’Union des Comores, actuellement présidée par Azali Assoumani. Il nous faudra aussi prendre des mesures opérationnelles pour restreindre l’immigration irrégulière, notamment en instaurant une véritable coordination entre nos forces de police terrestres,

visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte du député Philippe Gosselin. Ce texte a pour objet de prolonger une adaptation du droit de la nationalité aux conditions locales de Mayotte. En effet, le droit en vigueur depuis 2018 dans l’archipel mahorais impose qu’au moins l’un des parents d’un enfant étranger né sur le territoire séjourne depuis au moins trois mois en situation régulière pour que cet enfant puisse solliciter, en temps et en heure, l’acquisition de la nationalité française. Cette disposition est dérogatoire au droit de la nationalité en vigueur dans le reste du pays. Elle a été votée par le législateur afin de prendre en compte les particularités de Mayotte. La situation géographique de l’île, située dans le canal du Mozambique, a fait de ce territoire le point d’arrivée de flux migratoires importants en provenance des Comores et d’Afrique continentale. Or la perspective de l’acquisition de la nationalité française pour leurs descendants peut constituer une source de motivation non négligeable pour les arrivants, quand bien même elle ne serait qu’un critère parmi d’autres. Par ailleurs, comme cela a souvent été mentionné dans le cadre du débat sur la situation de Mayotte, la maternité de Mamoudzou est la plus active de France. Une part disproportionnée de la population de l’archipel est déjà composée de personnes de nationalité étrangère, souvent en situation irrégulière, irrégulière, y compris d’enfants nés de parents étrangers. Les circonstances matérielles dans lesquelles l’acquisition de la nationalité par le biais du mécanisme du droit du sol s’applique à Mayotte sont donc drastiquement différentes de celles qui prévalent en France métropolitaine, ou même dans les autres territoires ultramarins. C’est ce qui fonde une réponse législative différenciée, dont le principe fut approuvé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 septembre 2018. La présente proposition de loi, en allongeant le délai de séjour préalable des parents de trois mois à un an, s’inscrit donc dans la continuité de cette jurisprudence. Elle vise à diminuer l’attractivité du territoire mahorais et à limiter les flux migratoires, répondant ainsi aux attentes des Mahorais confrontés à la dégradation du contexte local. L’urgence est d’autant plus grande que le cyclone Chido a exacerbé l’ensemble des difficultés vécues sur le terrain. Répondre à cette attente tout en assurant la robustesse juridique du dispositif, tel était l’objet du texte que nous avons voté la semaine dernière, Depuis lors, notamment grâce à notre collègue rapporteur, Stéphane Le Rudulier, dont je salue le travail, la commission mixte paritaire a ouvert la voie à l’adoption d’une position commune des députés et des sénateurs. Le présent texte confirme en particulier le maintien à un an de la durée de séjour requise des parents – et non un

de la diversité des situations familiales, la commission mixte paritaire est parvenue à dégager un compromis permettant de requérir la résidence régulière des deux parents quand ceux ci sont connus, tout en adaptant le dispositif aux situations où un seul des parents est connu. Nous espérons que ce texte permettra d’offrir un commencement de réponse à l’une des multiples problématiques affectant le territoire mahorais, celle des flux migratoires. Il ne doit toutefois pas nous dispenser de réfléchir rapidement et efficacement à des solutions à l’ensemble des questions politiques, économiques, sociales et environnementales qui se posent à Mayotte, afin, en reprenant l’intitulé du rapport d’information élaboré en 2021 par notre commission des lois, de « conjurer le sentiment d’abandon des Mahorais ». Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains votera le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. La parole

réunis en commission mixte paritaire mardi dernier, députés et sénateurs sont parvenus à un accord pour renforcer les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte.

Pourtant, certains de nos collègues manifestent leur incompréhension face à la souffrance des Mahorais, las d’être privés de tout, et refusent de partager avec nous les étrangers arrivés à Mayotte, par péché dogmatique et en contradiction avec le mécanisme de solidarité institué entre pays de l’Union européenne. À défaut de mieux, nous avons retravaillé un mécanisme unique durcissant les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française à Mayotte, élaborée par le député Philippe Gosselin, ne nous satisfait pas. Le groupe RDSE souhaite rappeler son opposition nette à ce texte, qu’il s’agisse de la version adoptée à l’Assemblée nationale, largement anticonstitutionnelle, ou de celle adoptée par le Sénat, qui était certes plus raisonnable, mais tout aussi problématique sur le fond.

en CMP. Une sécurisation juridique relative aux familles monoparentales a certes été ajoutée, mais les arguments que nous avons avancés il y a quelques jours restent valables. Le texte issu de la commission mixte paritaire impose que les deux parents soient résidents réguliers depuis un an pour que leur enfant puisse revendiquer le droit du sol.

C’est même l’inverse : ces naissances ont augmenté de 14 %. Aujourd’hui, rien ne permet d’affirmer que le droit du sol est un facteur d’attractivité spécifique à Mayotte. De même, rien ne permet d’affirmer que durcir le droit du sol réduirait l’immigration.

commission, nous l’avons dit en séance et nous le redisons aujourd’hui : elle ne changera rien, si ce n’est qu’elle placera Mayotte encore plus en périphérie de la République. Le groupe RDSE votera contre. La parole

notre collègue Isabelle Florennes, vice présidente de la commission des lois et cheffe de file du groupe Union Centriste sur ce texte, ne pouvant être parmi nous ce matin, il me revient de vous faire part de la position de notre groupe sur les conclusions de la commission mixte paritaire. Chacun sait la situation de Mayotte, qui a été tragiquement mise en lumière par le passage du cyclone Chido, le 14 décembre dernier. Elle fait l’objet d’une attention régulière dans cette assemblée, qu’il s’agisse de l’accès à l’eau, de la précarité des services publics les plus fondamentaux ou de la pression migratoire intenable. Permettez moi de saluer, comme d’autres l’ont fait tout au long de l’examen de ce texte, l’engagement admirable des élus mahorais, qu’ils soient maires ou parlementaires. Ces lanceurs d’alerte vivent les difficultés de l’île au quotidien, ils les partagent avec la population. Il est donc de notre responsabilité de les écouter.

l’archipel sont d’origine étrangère et près d’un tiers d’entre eux seraient en situation irrégulière. Mes chers collègues, il n’est plus possible de nier que ces évolutions migratoires et démographiques pèsent massivement sur la vie quotidienne et les services publics mahorais. L’urgence sociale et migratoire qui règne à Mayotte nous oblige à agir en conscience.

Cette proposition de loi découle directement de la réflexion qui avait déjà conduit le législateur, il y a sept ans de cela, à adapter le régime du droit du sol à Mayotte en instaurant une condition supplémentaire relative à la régularité du séjour de l’un des parents au moment de la naissance de l’enfant. Les résultats étant loin d’être satisfaisants, il nous faut aller plus loin. Nos compatriotes mahorais nous le demandent ; nous les avons entendus. Nous renforçons ainsi les conditions d’accès à la nationalité, tout en veillant à garantir la constitutionnalité et l’applicabilité de ces nouvelles règles.

Pourtant, les Mahorais sont déjà discriminés : dans le cent unième département français, avant même les graves événements climatiques de décembre et janvier derniers, 77 % des habitants vivaient sous le seuil de pauvreté, 37 % d’entre eux étaient au chômage,

Pour quelle raison ? Aucun chiffre, aucune analyse ne démontre que les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte sont un facteur d’attractivité des flux migratoires. Si, depuis Si, depuis le durcissement législatif de 2018 en matière de droit du sol à Mayotte, le nombre de personnes devenues françaises a diminué, passant de 2 900 en 2018 à 860 en 2022, les flux migratoires se sont intensifiés dans le même Mes chers collègues, ne nous voilons pas la face : l’accès à la nationalité n’est pas le motif principal des migrations. Par ce texte, vous souhaitez dissuader les mères étrangères de venir donner vie à Mayotte. Mais ne soyons pas dupes, une personne étrangère ne consultera pas cette loi avant d’immigrer à Mayotte. La réalité de ces femmes est tout autre : c’est l’espoir d’une vie meilleure, le rêve de voir leurs enfants aller à l’école et la chance de pouvoir survivre en accouchant

on empêche délibérément ces personnes d’être en règle, pour les plonger toujours plus dans la précarité. Mes chers collègues, à Mayotte, le grand pays des droits de l’homme fait aujourd’hui le choix politique de se montrer hostile aux étrangers, en commençant par les enfants. Arrêtons d’utiliser Mayotte comme un laboratoire de dégradation des droits

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains. Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

Monsieur le président,

Le scrutin est ouvert.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.